Monsieur le président,

La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique est parvenue à l'adoption d'un texte commun.

de la lutte contre la covid et des mesures de coordination européenne, la situation actuelle, partout en Europe, suscite de vives inquiétudes. Partout, l'épidémie reprend, se développe ; partout, des mesures restrictives se mettent en place.

Face à la reprise de l'épidémie, nous devons reprendre nos travaux pour améliorer autant que possible cette coordination européenne. Il est normal que les mesures soient différenciées

au Conseil des affaires générales, auquel je participais, puis au Conseil européen, réunissant les chefs d'État et de gouvernement, pour harmoniser les seuils et les données scientifiques et sanitaires sur le fondement desquelles les mesures sont prises.

Sur le plan sanitaire, la question des vaccins a également été abordée à l'occasion du Conseil européen. Il faut souligner les avancées rapides de l'Union européenne pour assurer un travail commun.

Nous l'avons dit, nos pêcheurs ne valent pas moins que les pêcheurs britanniques, et notre priorité est de les défendre. Le maintien d'un accès durable, stable et réciproque aux eaux britanniques est évidemment notre priorité. Il importait de le rappeler clairement, parce que des critiques ou des doutes s'expriment

le 12 octobre dernier, l'ensemble des ministres concernés pour vérifier l'état de ces préparatifs, en vue de les accélérer ou de les compléter lorsque cela est nécessaire. Sur la question climatique, un premier débat

C'est la proposition de la Commission européenne ; le Parlement européen a voté un objectif plus ambitieux encore. Nous aurons l'occasion d'en reparler, mais il est impératif de conjuguer cette ambition avec une nécessaire équité.

de nos agriculteurs : oui au verdissement de la PAC, à condition que ses exigences s'appliquent à tous. Ces « écorégimes » constitueront au moins 20 % des paiements directs dans l'ensemble des États membres. discussion sur la PAC, un accord important a été obtenu par notre ministre de l'agriculture et de l'alimentation pour un soutien d'urgence à la viticulture française. Il vient compléter le plan présenté par le Premier ministre l'été

Les chances d'instaurer un partenariat étendu avec le Royaume-Uni après le 1 janvier 2021 s'amenuisent chaque jour davantage- votre ministre de tutelle, M. Le Drian,

Vous le savez, l'armée britannique est, avec l'armée française, celle qui compte en Europe ; membre du Conseil de sécurité des Nations unies, le Royaume-Uni doit rester associé à la défense de l'Europe -la géographie est têtue Le Sénat jouera tout son rôle pour conforter, sur le plan parlementaire, cette coopération. Ne laissons pas le Brexit ruiner ces dix années d'efforts

l'intégrité du marché intérieur. En Écosse, où 62 % des votes furent défavorables au Brexit lors du référendum de 2016, le camp des partisans de l'indépendance apparaît, désormais, majoritaire dans les sondages. Fragilisée elle aussi, l'Union européenne peine à s'affirmer comme puissance. À nos portes, la Turquie joue un rôle déstabilisateur, poussant sans vergogne ses pions de la Méditerranée orientale au nord-est syrien et au Haut-Karabakh, au mépris du droit international. Dimanche dernier, le candidat nationaliste Ersin Tatar, soutenu par la Turquie, a été élu président de l'autoproclamée République turque de Chypre-Nord. Il a battu le dirigeant sortant, qui était favorable à une réunification de l'île. Quelle sera la réaction européenne ? Quel corps prendra, concrètement, la fameuse « autonomie stratégique européenne » ? Les sanctions adoptées par le Conseil de l'Union européenne à la suite de l'affaire Navalny, tout comme les menaces de sanctions contre la Turquie lors du dernier Conseil européen,

la baisse des crédits du fonds européen de défense est un très mauvais signal, qui brouille les bonnes intentions affichées, y compris dans le domaine spatial. Face à l'affirmation des politiques de puissance au mépris du droit,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, si l'ordre du jour du Conseil européen de la semaine dernière était riche, avec notamment la question de la gestion de la crise sanitaire, ce sont en premier lieu les discussions relatives à la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne qui ont retenu l'attention de la commission de finances, compte tenu de son champ de compétences. Si ce Conseil européen était décrit comme le sommet de la dernière chance pour le Brexit, force est de constater qu'il a ressemblé aux précédents. Ce feuilleton, malheureusement désormais bien connu, reste inchangé les États membres ont manifesté leur union derrière le négociateur en chef, Michel Barnier, et ont constaté l'insuffisance des progrès accomplis jusqu'à présent. Dans une allocution prononcée à l'issue du Conseil européen, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a d'ailleurs soufflé sur les braises en regrettant que, après quarante-cinq années de participation britannique à l'Union européenne, cette dernière ne soit pas prête à accorder au Royaume-Uni un statut similaire à celui du Canada Toutefois, l'optimisme reste de rigueur, compte tenu de l'appel du Conseil européen à intensifier les négociations et de l'accord de Londres, annoncé ce soir, pour les reprendre. Ainsi, le Conseil européen n'a toujours pas tranché définitivement le sort du Brexit ; nous avons le sentiment d'assister à une partie d'échecs interminable. Les rebondissements de ces négociations font peser des incertitudes sur nos entreprises et sur de nombreux Français dont le quotidien est déjà bouleversé par la crise sanitaire actuelle. Dans ses conclusions, le Conseil européen appelle l'ensemble des parties prenantes, à tous les échelons, à intensifier leurs travaux pour se préparer à une éventuelle absence d'accord. Or le temps presse

notre assemblée examinera en séance publique le projet de loi de finances pour 2021. Les travaux ont déjà commencé en commission. Si les conséquences économiques de la crise sanitaire ont pu occulter, au cours des derniers mois, les débats sur les effets d'un sur l'économie française, maintenant que l'échéance est proche, les prévisions macroéconomiques ont nécessairement pu être affutées. Qu'en est-il concrètement ? Outre Outre les effets macroéconomiques, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne a des conséquences budgétaires immédiates sur le montant de la participation de la France au budget européen : celui-ci augmentera de 2,1 milliards d'euros

L'économie britannique a-t-elle réellement plus à craindre que la nôtre d'un retrait sans accord ? Les débats du Conseil européen ont également porté sur le changement climatique et, plus précisément, sur la proposition de la Commission européenne de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici à 2030. En ma qualité de rapporteur général de la commission des finances, mais aussi comme ancien rapporteur spécial des crédits de la mission « Écologie je salue la conduite d'une telle réflexion. À cet égard, la mobilisation du levier budgétaire semble indispensable. Dans cette perspective, en juillet dernier, le Conseil européen a invité la Commission à présenter une proposition visant à introduire une nouvelle ressource propre fondée sur un système révisé d'échange de quotas d'émission, en l'étendant éventuellement au transport maritime. Alors que les négociations relatives à la prochaine décision dite « ressources propres » de l'Union européenne sont en cours,

c'est un honneur pour moi, qui viens d'être élu président de la commission des affaires européennes, d'ouvrir ce débat consécutif à la réunion du Conseil européen des 15 et 16 octobre. Je tiens à rendre publiquement hommage à mon prédécesseur, Jean Bizet, qui a tant oeuvré pour toujours mieux faire entendre la voix du Sénat à Bruxelles et diffuser l'esprit européen au Sénat. Je l'en remercie et je tâcherai de poursuivre cette mission avec la même ardeur

Ce pays reste l'un des voisins les plus proches de l'Union européenne, il est fortement intégré commercialement à l'Union, et nous espérons tous construire avec lui une nouvelle relation privilégiée. Bien Bien sûr, le Royaume-Uni y a encore plus intérêt que nous : selon la Commission, il dépend de l'Union pour environ la moitié de son commerce de biens, alors que l'Union réalise 13 % de son commerce de biens avec lui. L'Union tient aussi un levier important avec le passeport financier, qu'elle peut décider unilatéralement d'octroyer, ou non, au Royaume-Uni. Le rapport de force est donc en notre faveur, mais nous sommes particulièrement soucieux pour nos pêcheurs, qui ont besoin de pouvoir travailler dans les eaux britanniques et dont l'activité est tributaire de l'issue de la négociation. Certains grands armements négocient déjà en sous-main des droits de pêche avec les Britanniques, voire rachètent des navires sous pavillon britannique. Or ces grandes manoeuvres sont hors de portée pour la pêche artisanale, qui fait vivre tant de familles sur nos côtes.

Et quand bien même un accord serait finalement conclu, comment être sûr qu'il sera respecté ? En effet, le projet de loi sur le marché intérieur britannique viole de manière flagrante l'accord de retrait conclu ensemble il y a seulement un an.

Mais nous entrons maintenant dans le vif du sujet : les États membres prennent la mesure de l'ampleur de l'effort à accomplir, et il n'est pas étonnant que les chefs d'État ou de gouvernement aient reporté à leur prochaine réunion de décembre la décision sur l'ampleur du relèvement de l'objectif de réduction des émissions de carbone.

Cette concession aux États aujourd'hui adeptes du charbon risque d'accroître la pression sur les autres, notamment sur la France. Aussi pouvons-nous légitimement nous interroger sur l'effort qui sera demandé à notre pays et sur ses conséquences pour nos industries et notre agriculture.

D'un côté, je me félicite de l'élan que semblent vouloir donner les chefs d'État ou de gouvernement à notre partenariat avec l'Afrique : c'est assurément le continent avec lequel l'Europe doit construire un avenir, en bâtissant sur un socle commun de valeurs partagées et en engageant des investissements substantiels dans les infrastructures, au service du développement durable. De l'autre, nous pouvons être inquiets de la frilosité du Conseil européen devant l'évolution de la situation en Biélorussie, au Haut-Karabakh ou encore en Méditerranée orientale, où la Russie et la Turquie multiplient les provocations. La diplomatie européenne doit absolument changer de braquet et permettre à l'Union européenne de se faire respecter sur la scène internationale. Comment la France peut-elle en convaincre ses partenaires ? je formulerai une observation conclusive. Alors qu'il doit normalement se réunir quatre fois par an, le Conseil européen s'est réuni deux fois pendant ce seul mois d'octobre : cette situation s'explique bien sûr par des impératifs sanitaires, mais elle traduit sans doute une évolution de fond dans la répartition des rôles entre les institutions de l'Union. Notre commission des affaires européennes en tiendra compte dans la réflexion qu'elle entend mener dans la perspective de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Cette conférence doit permettre aux Européens de se réapproprier la construction européenne : il est donc important qu'elle ait lieu, même si la pandémie a contraint de reporter son lancement, prévu en mai dernier.

Le vote du Parlement européen est une avancée inédite, mais elle ne paraît pas avoir été relayée par ce Conseil européen. Certes, le Conseil européen n'a pas tranché

d'ici à 2030, qui semble représenter le compromis déjà convenu à demi-mot. Manifestement, lors de ce Conseil européen, la ligne de la Commission européenne n'a pas été troublée.

le Sénat, chambre des territoires, doit aussi relayer les attentes des élus locaux. Ce sont eux, ce sont elles qui savent le mieux investir au plus près des citoyens pour traduire en actions concrètes les mesures de transition. Nous sommes donc très

de l'Union européenne, sur la gestion de la crise sanitaire, sur les pourparlers avec le Royaume-Uni dans la perspective du Brexit et sur la redéfinition de nos ambitions climatiques. L'Europe est là, et bien là

En Allemagne, l'épidémie connaît une nette accélération. En Espagne, des habitants sont appelés à rester chez eux. À Londres, et dans d'autres régions du Royaume-Uni, il est désormais interdit de recevoir chez soi des personnes extérieures au foyer. Une campagne de dépistage de tous les Slovaques de plus de dix ans va être lancée. Notre continent paie un lourd tribut, avec plus de 250 000 décès. Dans ce contexte de crise sanitaire, la gestion collective de la pandémie s'est nettement améliorée ces derniers mois. Le Conseil européen a appelé à ce que ces efforts conjoints des États membres se poursuivent, ce que nous ne pouvons qu'approuver. L'Union est aujourd'hui au rendez-vous et apparaît, dans ce domaine aussi, comme l'échelon pertinent d'intervention pour lutter contre la pandémie. Pour être plus efficaces encore, il nous faut en effet mener, au niveau européen, des actions coordonnées sur la base des meilleures données scientifiques collectées selon une méthodologie commune, de la recherche transfrontières des contacts, des stratégies de dépistage, de la reconnaissance mutuelle des tests, de la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l'Union européenne. À cet égard, je salue le travail du groupe Renew Europe, et plus particulièrement celui de notre collègue eurodéputée Véronique Trillet-Lenoir, qui a préfiguré l'adoption de recommandations par le Conseil des affaires générales du 13 octobre dernier, auquel vous avez participé, monsieur le secrétaire d'État. Nous saluons votre action décisive.

Alors que la Commission a présenté, il y a un mois, un plan visant à une réduction d'au moins 55 % d'ici à 2030 des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, la décision sera finalement prise en décembre, pour les cinq ans de l'accord de Paris. Il nous faudra être au rendez-vous. Je reprends les propos tenus récemment par l'eurodéputé Pierre Karleskind : « Ne soyons pas défaitistes face à l'immensité de ce qui est devant nous. » Alors, soyons ambitieux

Sénatrice du Finistère, je voudrais insister sur cette dernière pierre d'achoppement. Le Président de la République l'a rappelé avec force, jeudi dernier, comme il l'avait d'ailleurs déjà fait en début d'année : sur ce sujet, pas d'accord sans un bon compromis symétrique, pas d'accord sans visibilité.

sauf, peut-être, à ce qu'ils concluent des accords de pêche bilatéraux avec d'autres États, comme ils viennent de le faire avec la Norvège. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point, monsieur le secrétaire d'État ? Rappelons par ailleurs que, en cas de, le Royaume-Uni n'aura plus accès au système européen de l'énergie, ce qui lui coûtera plus d'un milliard d'euros par an. Londres se verra également réimposer des droits de douane et des quotas, fortement préjudiciables à son économie. Nos pêcheurs ont conscience que la situation ne sera pas la même à l'avenir qu'aujourd'hui. Il nous faudra les accompagner, et le soutien de l'Union européenne sera absolument nécessaire dans cette vient en effet s'ajouter aux conséquences économiques de la crise de la covid-19, ainsi qu'à des réglementations complexes et parfois contestées. Pas d'accord sans un bon compromis, pas d'accord sans visibilité, sans respect dans la durée : je l'ai dit,

nous nous félicitons de ce que les ministres européens de l'agriculture soient parvenus à un accord sur la nouvelle politique agricole commune, prévoyant des mesures environnementales fortes pour tous les États membres. La parole

la question des relations futures entre le Royaume-Uni et l'Union européenne était une nouvelle fois inscrite à l'ordre du jour du dernier Conseil européen. Vous l'avez indiqué, monsieur le secrétaire

Eu égard à la longueur de nos façades maritimes, l'économie côtière est fondamentale pour notre pays et la dynamique de nombreux territoires français en dépend : c'est une évidence.

je me réjouis, monsieur le secrétaire d'État, de votre engagement de faire figurer la pêche tout en haut de vos priorités. Il faut parvenir à un accord donnant-donnant. D'un côté de la Manche, nos pêcheurs doivent pouvoir accéder aux eaux territoriales britanniques pour que leur activité reste économiquement viable ; de l'autre, nos amis Britanniques ont besoin de pouvoir accéder au marché européen pour écouler leurs produits : faut-il le leur rappeler ? Dans ces conditions, il faut refuser l'annualisation de l'accès aux eaux britanniques. Cette formule est même un non-sens économique, en ce qu'elle interdirait tout investissement, faute de visibilité d'une année sur l'autre. Elle ouvrirait la porte à une insécurité économique insoutenable pour nos pêcheurs. La pêche est un métier difficile, parfois dangereux, mais exercé avec passion. Je vous laisse imaginer le chaos qu'induirait la conclusion d'un mauvais accord. La France, avec les huit autres États membres concernés, doit tenir le cap d'une répartition juste des quotas d'espèces et d'un accès aux eaux réciproque et équitable.

Pour lutter contre le changement climatique, l'agriculture et la forêt représentent une partie de la solution. Trop souvent, l'agriculture est perçue comme une activité émettrice de gaz à effet de serre ; elle l'est,

C'est pourquoi j'adhère à cette nouvelle ambition formulée pour la PAC, et, dans ce cadre, je soutiens la position du Gouvernement de porter à 30 % le niveau des aides directes conditionnées au respect des mesures en faveur de l'écologie.

de ces stratégies, monsieur le secrétaire d'État, où en est le travail de la Commission sur l'élaboration d'un étiquetage nutritionnel harmonisé et d'un cadre pour l'étiquetage des denrées alimentaires durables couvrant les aspects nutritionnels, climatiques, environnementaux et sociaux des produits alimentaires C'est aussi parce que l'agriculture a un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique que nous devons accepter le verdissement de la politique agricole commune. Alors oui, comme le souligne le Conseil européen dans ses conclusions,

de covid-19. Dans ce contexte sanitaire, le sujet ne pouvait être évité, bien que l'Union européenne n'ait, pour l'heure, aucune compétence en matière de santé. Les questions relatives au changement climatique, ainsi

d'autant que, dimanche dernier, les deux camps se sont accusés mutuellement d'avoir violé une nouvelle trêve humanitaire, à peine une semaine après un premier cessez-le-feu, conclu mais jamais respecté. Les combats se poursuivent donc sur ce territoire où l'on compte déjà des centaines de morts et des dizaines, voire des centaines, de milliers de personnes affectées par le conflit, directement ou indirectement, et jetées sur les routes de l'exil. Mes chers collègues, il ne s'agit pas d'un fait mineur : la paix est menacée aux portes de l'Europe, et j'aimerais dire ici toute ma solidarité aux familles endeuillées, qui continuent de fuir les bombardements, laissant tout derrière elles. Compte tenu de ses relations avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais aussi de son implication dans le groupe de Minsk, la France ne peut que s'inquiéter de ces évolutions périlleuses qui éloignent la perspective d'une résolution pacifique du conflit. À quand une reconnaissance officielle par la France de la république d'Artsakh, en lieu et place de la représentation permanente installée en 1998 ? À quand une reconnaissance par l'Union européenne, qui a fait du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes un principe fondamental ? Nous estimons qu'une telle reconnaissance officielle constitue aujourd'hui le seul moyen de parvenir à une paix durable dans une zone instable depuis le fragile cessez-le-feu de mai 1994.

avec l'Azerbaïdjan sur la révision de l'accord de coopération de 1996 ? Comment comprendre les récentes déclarations de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, selon lesquelles, sur les dossiers chypriote, libyen libyen et artsakhi, des sanctions contre Ankara sont « prêtes et peuvent être utilisées immédiatement » ? Par ailleurs, dans le cadre offert par le groupe de Minsk, le strict respect des principes de Madrid de 2007 permettrait d'organiser à la fois un processus d'autodétermination sécurisé par une opération de maintien de la paix et le retour de plus d'un million de déplacés artsakhis, arméniens et azéris. Dans l'urgence de la situation, une question simple se pose : quelle est l'approche de l'Union européenne pour que les cessez-le-feu soient enfin respectés, notamment afin que puissent être dispensés les soins et l'aide aux populations civiles ? Selon nous, l'assistance civile, l'appui concret à la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu et la reconnaissance officielle de la république d'Artsakh sont aujourd'hui les seules solutions pour aboutir à une résolution pérenne du conflit. Il est regrettable que l'Union européenne ne soit pas à la hauteur de l'enjeu, eu égard à la catastrophe humanitaire qui se déroule devant nos yeux. La parole

J'ai déjà eu l'occasion de le souligner, le vote historique intervenu en la matière au Parlement européen le 6 octobre dernier, a fixé pour 2030 un objectif de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre de 60 par rapport à 1990, afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050. D'aucuns jugent cet objectif irréaliste ; d'autres s'en réjouissent.

en vue d'unir nos forces sur la scène mondiale pour continuer à faire progresser la cause de la lutte contre le changement climatique. Cela est primordial, car, qu'il s'agisse de la crise sanitaire que nous traversons ou de la

Septembre 2020 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde ; il y a urgence. Le climat de notre planète s'est déjà réchauffé de plus de 1 degré et il gagne encore, en moyenne, 0,2 degré par décennie depuis la fin des années 1970 ; il y a urgence. Les climatologues relèvent que les événements climatiques extrêmes sont devenus une nouvelle normalité. « Désormais, aucun endroit ni aucun d'entre nous n'est à l'abri du changement climatique nous prévient le climatologue américain Michael Mann, de l'université de Pennsylvanie ; il y a urgence. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable s'implique et s'impliquera dans la définition des orientations qui seront prises lors du prochain Conseil européen ; elle apportera toute sa part à l'élaboration de solutions en vue de réduire l'empreinte environnementale et climatique de notre économie.

Nous continuerons à combler ces angles morts de nos politiques publiques, en étant force de proposition pour une transition durable de notre économie. La parole

déjà mis à mal par le gouvernement britannique, en particulier pour assurer le respect des droits des Britanniques qui vivent dans l'Union européenne et des ressortissants de l'Union européenne qui continueront à vivre au

Vous nous direz également comment vous envisagez de sortir de la problématique de l'État de droit. Personne n'est parfait dans l'Union, beaucoup d'États se voient infliger des condamnations par la Cour de justice de l'Union européenne. Quels critères objectifs retenir

Concernant les relations extérieures, je pourrais reprendre mot pour mot les propos de notre collègue Jérémy Bacchi sur l'agression azérie au Haut-Karabakh.

revenir sur l'un point qui y figurait : la lutte contre le changement climatique. Atteindre la neutralité carbone en 2050, comme s'y est engagée l'Union européenne dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, nécessite de revoir à la hausse notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

Il est un fait que si nous sommes souvent très volontaires quand il s'agit de nous fixer des objectifs ambitieux, nous sommes un peu moins performants lorsqu'il s'agit de les tenir. Je rappelle, pour ne citer que l'exemple français, que notre pays n'est pas à la hauteur des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, engagements qui ont été traduits au plan national par la stratégie bas-carbone. nos émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 0,9 % l'année dernière, alors qu'elles auraient dû baisser de 1,5 %. Nous sommes donc loin de ces objectifs, sachant que, à partir de 2024, cette baisse est supposée atteindre 3,2 % par an. Il nous faut donc impérativement accélérer le rythme de réduction de nos émissions, comme le Haut Conseil pour le climat le souligne d'ailleurs dans son rapport annuel publié le mois dernier. Dans le cadre du plan d'investissements du Pacte vert pour l'Europe et du plan de relance européen, qui sera financé par de la dette commune, l'Union européenne entend mobiliser des moyens considérables

Il est prévu qu'au moins 30 % de cette capacité financière soit consacrée aux dépenses liées au climat, les autres dépenses devant respecter le principe consistant à ne pas nuire à l'environnement. Au regard des défis auxquels notre continent fait face et des besoins colossaux en l'investissement, nombreux sont ceux qui considèrent que ce montant est insuffisant. De même, plusieurs questions se posent s'agissant de l'utilisation de ces moyens : selon quels critères seront-ils utilisés ? Comment distinguer des projets qui concourent réellement à cette transition ? Comment s'assurer que cette manne financière viendra bien financer des investissements verts ? Et à quel rythme pourra-t-elle être débloquée ? Nous sommes par ailleurs en attente, monsieur le secrétaire d'État, d'une véritable stratégie européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports. En effet, les stratégies relatives à la transition agricole et à la transition énergétique ont été récemment publiées. Les transports sont, au niveau européen, le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. En France, il s'agit même du premier secteur émetteur, qui contribue à près de 30 % de nos émissions totales, et c'est le seul secteur dont les émissions, au lieu de diminuer, ont augmenté depuis 1990. La majorité de ces émissions sont liées au transport routier. Comme le souligne la Commission européenne dans sa communication du 17 septembre sur les ambitions de l'Europe en matière de climat pour 2030, ce secteur pourrait enregistrer une diminution de ses émissions d'environ 20 % seulement entre 2015 et 2030, ce qui nécessite qu'il fasse l'objet d'une attention accrue. Or, en dehors de quelques mesures prises par l'Union européenne, par exemple en matière de normes d'émissions des véhicules particuliers et des poids lourds, on peine à trouver au niveau européen un plan d'action ambitieux en faveur de la décarbonation des transports. Pourtant, les investissements réalisés ne manquent pas. À quand, monsieur le secrétaire d'État, un grand plan d'investissement européen en faveur des transports publics et des transports ferroviaires, fluviaux et maritimes ? C'est peu dire que la stratégie pour une mobilité durable et intelligente que la Commission européenne entend bâtir ces prochains mois est importante. Elle devrait permettre d'aller plus loin dans le soutien à la conversion du parc automobile, au développement des carburants alternatifs, au développement des transports publics et, plus généralement, au report modal. En ce qui concerne les transports maritimes, un mouvement de verdissement est d'ores et déjà engagé, au travers notamment du développement de navires à propulsion au gaz naturel liquéfié, ou GNL. Pour autant, de gros efforts restent à fournir pour réduire les importantes émissions de CO2, d'oxyde d'azote, d'oxyde de soufre et de particules fines des navires et développer les carburants alternatifs. La Commission européenne et le Parlement souhaitent par ailleurs inclure le transport maritime au sein du marché carbone- Jean-François Husson l'a souligné précédemment. Quelle est la position de la France sur cette proposition, monsieur le secrétaire En matière de transport aérien, les engagements pris avant la crise sanitaire continuent pour l'heure d'être suivis par les compagnies aériennes et les aéroports. En juin 2019, plus de 200 aéroports européens ont signé la résolution du Conseil international des aéroports, ou ou ACI, s'engageant dans une feuille de route visant à atteindre l'objectif zéro émission nette de CO2 au plus tard en 2050. Airbus s'est fixé comme objectif d'être le premier constructeur à proposer, en 2035, l'avion à hydrogène. Néanmoins, le secteur mettra des années à retrouver son activité de 2019, et le choc économique lié à la crise sanitaire risque que de remettre en question ces objectifs. Quelle politique européenne est-elle envisagée pour soutenir les objectifs de décarbonation

parmi les sujets traités dans le cadre de ce Conseil européen, j'évoquerai deux points qui sont complémentaires de l'intervention de mon collègue Jean-François Longeot, président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du développement durable : les négociations entre Londres et Bruxelles et les évolutions dans la gestion de la crise sanitaire mondiale que nous vivons. Depuis que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne, les pourparlers entre Londres et Bruxelles pour un accord de libre-échange qui entrerait en vigueur à la fin de la période de transition patinent, et l'échéance se rapproche dangereusement.

par l'absence de quotas de pêche partagés et par le retour possible de nouveaux conflits d'usage entre les flottilles françaises, belges et néerlandaises dans la zone de pêche largement amputée au niveau de la Manche. Très dépendante de la future négociation, la filière pêche française sera lourdement menacée par une absence de traité et d'accès réciproque dans les eaux territoriales. Entre 2011 et 2015, quelque 98 000 tonnes de poissons ont été pêchées chaque année dans les eaux territoriales britanniques, entraînant 171 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2 566 emplois directs. Nous sommes en vision englober la englober la pêche dans un accord global de libre-échange reste un réel contrepoids dans les négociations. Quelque trente ports français sont concernés par cette dépendance. Permettez-moi, pour illustrer mon propos, de prendre l'exemple de mon territoire, les Hauts-de-France, deuxième région la plus fortement touchée. Le port de Boulogne-sur-Mer est le premier port de pêche français en termes de tonnage- 36 000 tonnes par an. On y traite 360 000 tonnes de produits de la mer chaque année. Sa logistique d'approvisionnement et de distribution et sa capacité frigorifique sont sans équivalent pour la filière. Boulogne-sur-Mer est une plateforme logistique agroalimentaire leader en France Ne devrions-nous pas mieux anticiper la crise par plusieurs dispositifs, par exemple en assouplissant le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, afin de pouvoir l'utiliser comme un fonds d'urgence de soutien du secteur, ou en mettant en place un plan stratégique pour l'avenir de la pêche européenne,

assure chaque année le transport de 10 millions de voyageurs, mais aussi de 44 millions de tonnes de marchandises sur la ligne de ferry Calais-Douvres. C'est un un poumon économique pour notre territoire. L'Union européenne doit se doter d'un accord de libre-échange ambitieux. S'il souhaite maintenir des relations commerciales sans quotas ni droits de douane, le Royaume-Uni doit s'engager à actualiser ses règles

d'aborder un dossier tout particulier : la concession franco-britannique Eurotunnel, filiale de Getlink, qui assure 26 % des échanges entre le Royaume-Uni et le continent européen, soit un peu plus de 138 milliards d'euros de marchandises et 21 millions de passagers par an. L'Union européenne a encouragé la France à négocier un avenant au traité de Canterbury, pour faire en sorte que le tunnel reste sous l'égide du droit européen et de la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne en cas de litige. Qu'en est-il de cette concertation,

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le constat du réchauffement climatique et de la destruction des espaces naturels est réel. Les citoyens européens nous interpellent, nous, les élus, sur la nécessité d'agir pour la planète, pour l'humanité et pour les générations à venir. L'Union européenne a compris la nécessité de bâtir un modèle économique viable en tenant compte de l'urgence climatique. Pourtant, l'action européenne en faveur du climat a été évoquée au Conseil européen des 15 et 16 octobre sans que soit arrêtée de position concernant la révision de l'objectif de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon de 2030, objectif qui s'intègre dans la stratégie de l'Union européenne en vue d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2050.

Les conclusions des 15 et 16 octobre confirment bien la volonté de convenir lors du Conseil européen de décembre, à la fois d'un nouvel objectif de réduction des émissions pour 2030 plus ambitieux, mais aussi de l'actualisation de la contribution déterminée au niveau national de l'Union européenne, qui sera adressée aux parties à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique. Bien que la cible finale pour l'horizon 2030 ne soit pas précisée, les conclusions se réfèrent à la proposition présentée par la Commission européenne de réduire d'au moins 55 % les réductions d'émissions d'ici à 2030. est donc la suivante, monsieur le secrétaire d'État : cela signifie-t-il que, dès aujourd'hui, la position adoptée par le Parlement européen le 6 octobre à une courte majorité de relever cet objectif à 60 % est jugée hors de portée, donc exclue pour le Conseil européen ? Ce nouvel objectif pour 2030 sera atteint collectivement par l'Union européenne, ce qui implique des différences et une solidarité entre les États dans une logique d'équité et de maîtrise des coûts.

souhaite saluer cette décision -a appelé la Commission à mener des consultations approfondies avec les États membres, afin d'évaluer les situations spécifiques et de fournir davantage d'informations sur les répercussions de ce nouvel objectif à l'échelon des États membres. À ce stade, monsieur le secrétaire d'État, je souhaiterais que vous nous éclairiez sur l'état des réflexions et des rapports de force au sein du Conseil européen, à la fois sur l'ambition révisée, mais aussi sur le niveau acceptable ou souhaitable de solidarité entre les États pour y parvenir. Compte tenu des premiers échanges intervenus avec la Commission, pouvez-vous également d'ores et déjà nous éclairer sur l'impact prévisionnel d'un tel rehaussement pour la France ? Enfin, les conclusions du Conseil des 15 et 16 octobre évoquent la nécessité de prévenir le risque de fuite carbone- vous l'avez évoqué. C'est un sujet auquel le Sénat est particulièrement sensible. Il est essentiel de mettre en place rapidement un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, afin de préserver des conditions équitables de concurrence entre les entreprises européennes et les autres, mais aussi de répondre à cet enjeu de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui a une portée mondiale. L'Europe ne doit pas se montrer naïve en la matière. Ces débats prouvent bien, comme l'avait affirmé le Sénat dans son avis motivé relatif à la loi européenne sur le climat, que la définition de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre n'est pas un élément technique ni mécanique elle revêt un caractère éminemment politique et doit être pleinement acceptée par les États membres pour être mise en oeuvre avec succès. Les enjeux d'une telle décision sont lourds en termes économiques et sociaux, technologiques et industriels, mais aussi en termes d'aménagement du territoire dans chacun des États membres ; il ne faut pas se le cacher. Je me félicite donc de ce que la dernière position de compromis sur la loi européenne sur le climat, présentée par la présidence allemande en vue du Conseil « Environnement » du 23 octobre, écarte la voie du recours aux actes délégués entre 2030 et 2050 et retienne en contrepartie le principe d'un objectif intermédiaire à l'horizon de 2040. Tel était le point dur de l'avis motivé du Sénat. est toutefois de parvenir à mettre en oeuvre de manière concrète et efficace les instruments du cadre financier pluriannuel et du plan de relance, notamment en vue d'accompagner les défis économiques, sociaux et territoriaux de la lutte contre le changement climatique dans un contexte économique profondément dégradé La lutte contre le changement climatique est l'une des matrices structurantes de ce nouveau cadre financier pluriannuel et du plan de relance. Plus l'Europe prend du retard dans leur mise en oeuvre, plus il lui sera difficile d'atteindre un objectif rehaussé de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions satisfaisantes. La parole

Dans le contexte actuel, la question qui me semble la plus fondamentale est la suivante : comment faire de l'Union européenne un outil stratégique pour écrire la prochaine page de la mondialisation ? L'Europe peut saisir cette opportunité pour redonner un sens à la mondialisation.

vise un double objectif : économique, par la restauration de la compétitivité de nos entreprises et de nos agriculteurs soumis à des normes beaucoup plus exigeantes que leurs partenaires commerciaux ; et écologique, par la taxation des produits provenant des pays s'affranchissant de toute réglementation environnementale. Je crois à l'échange, à la force de nos entreprises, à la compétence de nos salariés et de nos agriculteurs et à l'excellence de leur savoir-faire. Mais, pour que cette liberté d'échanger ait un sens, il faut que les règles soient les mêmes pour tous et que nous remettions de l'équité et de la réciprocité dans les échanges internationaux. Pour que l'écologie et la lutte contre le dérèglement climatique soient non pas dogmatiques, mais pragmatiques et durables, pour qu'elles protègent nos emplois, la mise en place de cette barrière écologique semble essentielle. Nous avons besoin d'actes réels. Trop souvent, les politiques publiques environnementales peuvent sembler inconsistantes. C'est d'autant plus vrai lorsqu'elles sont européennes : les objectifs sont soit fixés à très long terme et ne nous engagent pas réellement, soit fixés à court terme et irréalistes, discréditant ainsi la parole publique. En matière de climat et d'énergie, nos objectifs doivent être réalisables et ils doivent respecter une règle simple : arrêtons de créer des usines à gaz trop sophistiquées. Conformément aux objectifs de l'accord de Paris, l'Europe- tout le monde en est d'accord -doit s'engager sur un objectif de neutralité carbone ou neutralité climatique à l'horizon 2050. La Commission a estimé qu'il fallait rehausser les objectifs climatiques européens pour 2030, car les politiques actuelles ne permettront de de réduire les émissions de gaz à effet de serre que de 60 % d'ici 2050. Mais quelle ambition et quelles mesures concrètes ? Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite également évoquer le sujet de l'agriculture, si stratégique pour

des mesures législatives pour une diminution de l'utilisation des pesticides, des mesures favorisant l'augmentation des surfaces consacrées à l'agriculture biologique et des actions visant à aider les consommateurs à opter pour une alimentation saine et durable.

créés, afin d'éviter les distorsions de concurrence pour nos agriculteurs. Sachez que nous serons particulièrement vigilants sur ce point, car nous avons besoin de l'agriculture pour l'écologie de l'agriculture pour l'écologie : les agriculteurs concourent largement à la diversité biologique par l'élevage, par la variété des cultures et par l'entretien de nos paysages. Nos agriculteurs ont besoin du soutien de l'Europe, Enfin, dans tous les pays européens nous devons bâtir des approches territoriales et proposer une adaptation des politiques publiques à la lutte contre le changement climatique. Il faut donc passer à l'action dans les territoires et faciliter le dialogue entre l'État, les

plus fermes dans la défense des intérêts de pêcheurs qui en dépendent directement. Je rappelle que, au total, sur la façade nord-est du pays, ce sont entre 25 % et 30 % de la pêche qui s'effectuent directement dans les eaux britanniques aujourd'hui.

le nôtre. Si l'on prend la filière halieutique au sens large, en y incluant la transformation, il y a un besoin britannique presque vital, notamment à court terme, d'accéder

À cet égard, je crois que l'activisme climatique ou la diplomatie climatique européenne a été efficace, puisque la Chine, par exemple, vient d'endosser une cible en matière de neutralité carbone, qui n'est certes pas l'échéance de 2050, mais qui est 2060, ce qui n'est pas neutre ou anodin.

me semble-t-il, le Conseil européen a demandé à la Commission européenne de détailler cette étude d'impact

sans une politique agricole commune bien financée au niveau européen. En effet, celle-ci contribuera très largement à l'accomplissement de cette ambition, dans les conditions de verdissement que j'évoquais dans mon intervention liminaire, à savoir les « écorégimes » obligatoires négociés par Julien Denormandie, qui, je l'espère, seront confirmés, voire renforcés

notamment pour l'Arménie, est que les hostilités cessent. En tant que coprésidente du groupe de Minsk- le Président de la République s'est entretenu à plusieurs reprises avec le président Trump et le président Poutine,

au tunnel sous la Manche. En effet, le traité de Canterbury ne suffit pas : certaines règles en matière de sécurité ou les licences des conducteurs de train dépendent directement des règlements ferroviaires européens. Il faut donc trouver un équivalent, que la France va négocier avec le Royaume-Uni. Si nous n'aboutissions pas à un accord,

de contingence unilatérales et symétriques, pour garantir que, en tout état de cause, le tunnel fonctionne dans des conditions de sécurité communes et respectées. Je crois avoir répondu aux questions de Mme de Cidrac sur le climat. J'ajouterai un dernier point au sujet des outils d'accompagnement

internationaux qui ne respectent pas nos exigences minimales en matière sanitaire et environnementale. Je pense évidemment, vous l'aurez compris, à l'accord sur le Mercosur, qui a justifié une position de rejet et de fermeté de la France.